en date du 10 mars 2021, le Gouvernement demande de modifier l'ordre du jour des jeudis 1 et 8 avril 2021. Concernant l'ordre du jour du jeudi 1 avril 2021, le Gouvernement demande de compléter l'ordre du jour du matin

demande également l'inscription, l'après-midi, sous réserve de sa transmission, avant la suite du projet de loi confortant le respect des principes de la République, de la nouvelle lecture de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

Concernant l'ordre du jour du jeudi 8 avril 2021, le Gouvernement demande l'inscription, le matin, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi rénovant la gouvernance du service public d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe ou de sa nouvelle lecture.

Paulette Guinchard-Kunstler, a décidé de finir sa vie en Suisse, dans un pays qui pouvait l'accueillir. Que nous dit ce choix intime de la situation qui est la nôtre, en France ?

Le premier à l'avoir soulevé a été Henri Caillavet, en 1978. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) a été créée en 1980.

et placée dans une situation personnelle extrêmement douloureuse, elle a évolué, s'est tournée vers le monde médical et a découvert que la loi Claeys-Leonetti ne pouvait lui être d'aucune aide.

peut-être plus fortes que celles que connaît la France. Par ailleurs, et c'est toute la particularité de ce sujet, nos compatriotes sont massivement favorables

le recours par des Français à l'euthanasie et au suicide assisté est une réalité, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur même de nos frontières. Plusieurs d'entre eux se rendent chaque année en Belgique pour bénéficier d'une euthanasie ou en Suisse pour obtenir une assistance au suicide.

Tout comme pour l'écrivaine Anne Bert, contrainte de solliciter en 2017 une euthanasie en Belgique, l'ultime recours de Paulette Guinchard-Kunstler nous renvoie à la détresse et à l'angoisse existentielle de nombre de nos concitoyens, que notre législation en matière de fin de vie ne permet pas d'apaiser. Gardons également à l'esprit une autre réalité, impossible à objectiver : le nombre important de malades atteints d'une affection grave et incurable qui n'ont ni les moyens ni la force de se rendre en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, mais qui ne peuvent pas non plus bénéficier des dispositifs d'accompagnement de la fin de vie institués par la loi Claeys-Leonetti de 2016. À ces départs à l'étranger s'ajoutent les euthanasies dites clandestines réalisées sur notre territoire : comme l'a rappelé en 2018 le Conseil économique, social et environnemental, entre 2 000 et 4 000 décès annuels résulteraient d'une euthanasie active pratiquée par des professionnels de santé en dépit de son interdiction par la loi. Avant d'entrer dans le détail des insuffisances de la loi en vigueur, j'insisterai sur le devoir de modestie auquel nous sommes tous tenus, élus comme professionnels de santé, lorsqu'il s'agit d'aborder une question aussi délicate que la fin de vie. Personne ne peut se prévaloir de certitudes sur la manière dont une personne affectée par une maladie incurable appréhende les derniers jours de sa vie et la conception qu'elle se fait d'une fin de vie digne. Nous devons donc nous garder de juger les choix, très personnels et propres à chaque situation, qui sont faits en fin de vie. Cinq ans après l'adoption de la loi Claeys-Leonetti, le bilan est mitigé. Si cette loi a permis des avancées indéniables grâce au caractère contraignant des directives anticipées et à la désignation de la personne de confiance, son application reste insatisfaisante. son dispositif principal, la sédation profonde et continue, ne permet pas de répondre à certaines demandes d'accompagnement de la fin de vie, pourtant parfaitement entendables, au regard de la souffrance du patient. En 2018, l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) a pointé en particulier l'absence de registre national des directives anticipées et le défaut de traçabilité des décisions d'arrêt des traitements et d'administration de la sédation profonde et continue jusqu'au décès.

Monsieur le ministre, quand le Gouvernement compte-t-il autoriser la dispensation du Midazolam en ville, alors que la Haute Autorité de santé la préconise depuis le En dépit des progrès indéniables qu'elle a permis, la loi de 2016 présente des limites qui interrogent le devoir d'humanité, de solidarité et de compassion incombant incombant à notre société. Tout d'abord, en circonscrivant la possibilité de bénéficier de la sédation profonde et continue jusqu'au décès à des situations soit d'imminence de la mort, soit d'obstination déraisonnable pour les personnes hors d'état d'exprimer leur volonté, ce texte ne laisse finalement encore que que peu de place à la volonté du patient. L'appréciation du caractère insupportable de la souffrance par le médecin semble rester prépondérante dans bien des cas. La souffrance existentielle du patient demeure ainsi difficilement appréhendée par les équipes soignantes, qui restent attachées à une objectivation de la souffrance sur la base de symptômes cliniques. Ensuite, les critères de l'obstination déraisonnable, de la souffrance réfractaire aux traitements et de l'engagement du pronostic vital à court terme paraissent peu pertinents dans un certain nombre de situations qui, bien que limitées dans leur nombre, sont à l'origine d'une souffrance considérable pour les personnes concernées. Je pense à des maladies neurodégénératives particulièrement graves, telles que la maladie de Charcot, pour lesquelles l'évolution gravement incapacitante de la maladie est la source d'une angoisse existentielle difficilement soutenable.

chroniques. Les éventuels conflits entre la famille et l'équipe soignante dans l'interprétation de la loi rendent alors difficile l'établissement de la volonté du patient par le médecin. Face à ces situations qui exigent de concilier respect du libre arbitre et protection de la vulnérabilité, notre législation doit rester attentive aux attentes de l'opinion publique, ainsi qu'aux évolutions

96 % des Français interrogés se sont déclarés favorables à la reconnaissance et à l'encadrement d'un droit à l'euthanasie. Par ailleurs, plusieurs pays étrangers reconnaissent un droit à l'aide active à mourir, dans le souci de mieux respecter l'autonomie de la personne et son souhait de mourir dans des conditions qu'elle juge dignes : les pays du Benelux bien sûr, mais aussi la Suisse, le Canada, plusieurs États aux États-Unis et en Australie, plus récemment la Nouvelle-Zélande et le Portugal. L'Espagne ce droit. Dans ces conditions, la France sera bientôt frontalière de quatre pays autorisant une ou plusieurs modalités de l'aide active à mourir. Ces législations étrangères peuvent apporter aux patients un surplus d'apaisement psychologique dans l'appréhension de leur fin de vie, sans pour autant les conduire à systématiquement passer à l'acte, tout en garantissant la traçabilité et le contrôle de ces situations. Dans ces conditions, la proposition de loi dont Marie-Pierre de La Gontrie est la première signataire consacre le droit à une fin de vie digne, en y incluant le droit à bénéficier de l'aide active à mourir, mise en oeuvre par le suicide médicalement assisté ou par l'euthanasie. Elle définit également des critères exigeants qui conditionneront le bénéfice de cette aide active à mourir. Dans le respect du libre arbitre du patient, ces critères accordent une place déterminante à l'appréciation que celui-ci fait de sa situation, du caractère insupportable de sa souffrance physique ou psychique ou du caractère indigne de son état de dépendance. dans les législations des pays du Benelux, la mise en oeuvre des aides actives à mourir fera, en outre, l'objet d'un contrôle par une commission nationale qui en assurera la traçabilité. La proposition de loi ne se cantonne pas à la reconnaissance de l'aide active à mourir. Elle veille également à garantir le respect des volontés de la personne ayant perdu leur capacité, en rénovant notamment le cadre juridique applicable aux directives anticipées pour améliorer leur développement et renforcer leur caractère contraignant. Enfin, dans le souci d'apporter une réponse globale au « mal mourir » en France, la proposition de loi prévoit de rendre effectif un droit universel à l'accès aux soins palliatifs et à un accompagnement en tout point du territoire

Il nous ramène tous à ce que nous sommes fondamentalement : des êtres marqués par la finitude. Parler de la fin de vie et de la façon dont la société la regarde, plus ou moins en face, plus ou moins de biais, c'est placer au

Comme aide-soignant en Ehpad, comme médecin neurologue et, à ce titre, confronté à des maladies parfois aiguës, parfois chroniques, très dures, j'ai assisté de près à ces moments où un résident, un patient, est confronté à l'imminence de sa mort. Loin des convictions tranchées et des positions inébranlables, ces moments représentent toujours une épreuve de vérité, avec ses doutes, ses hésitations, ses angoisses et ses craintes souvent, sa sérénité parfois. Dans le débat qui s'engage, je sais que nous serons à la hauteur de ces doutes. Commençons par regarder ce que la France prévoit d'ores et déjà en matière de fin de vie. Il y a très précisément cinq ans a été votée dans cet hémicycle la loi

Elle a notamment réaffirmé le droit du malade à l'arrêt de tout traitement. Elle a rendu contraignantes les directives anticipées pour les médecins. Répond-elle pour autant à toutes les situations individuelles ? Peut-être pas. En cet instant, j'ai moi aussi une pensée émue pour Paulette Guinchard-Kunstler, femme engagée, militante infatigable, ancienne secrétaire d'État aux personnes âgées, qui vient de nous quitter dans les conditions qui ont été rappelées. Il me semble néanmoins, comme à de nombreux observateurs, notamment le Comité consultatif national d'éthique (CNCE), qui a rendu un avis sur ce thème en 2020, que la loi actuelle pose en droit un cadre qui permet de résoudre l'immense majorité des situations difficiles que peuvent vivre les patients, leurs familles et, parfois, il faut le rappeler,

aux professionnels de santé, aux professionnels des soins palliatifs, aux accompagnants et aux bénévoles qui travaillent dans ces services et, bien entendu, à tous les Français. Pour ne donner qu'un exemple, qui donne une idée du chemin à parcourir, je

Il y a donc du travail, je le concède, et la crise sanitaire nous a sans doute fait perdre un temps précieux, tout autant qu'elle aura mis en lumière nos propres insuffisances. Durant la crise sanitaire, j'ai été amené à autoriser

alors secoué une partie de la société et les réactions parfois extrêmement violentes que j'ai pu essuyer de la part d'une partie de la population qui considérait que soulager des souffrances devenues insupportables et irrémédiables s'apparentait à une forme de je ne sais quel génocide programmé. La situation n'est pas si simple. Avant de soutenir que la population

Assurer la mise en oeuvre concrète et réelle du cadre existant constitue en revanche un travail urgent, sur lequel le Gouvernement vous propose d'accélérer et dont la tâche m'incombe en tant que ministre chargé des questions de santé. Je m'attelle d'ores et déjà à ce travail : je tiens à vous annoncer aujourd'hui le lancement, à compter du mois d'avril prochain, d'un nouveau plan national de développement des soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de vie. Il s'agira du cinquième plan national, le précédent s'étant il est vrai interrompu en 2019. Je confierai à mes confrères Olivier Mermet et Bruno Richard, unanimement reconnus pour leur implication sur le sujet, le soin de copiloter ce nouveau plan national triennal. Mieux faire connaître la loi actuelle aux professionnels et aux accompagnants sera l'un des fils conducteurs de ce plan, qui sera largement détaillé au cours des prochaines assises de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs au mois de mai prochain. Nous inscrirons dans ce plan la nécessité d'améliorer la formation initiale et continue de l'ensemble des professionnels de santé sur la thématique de la fin de vie. Avec Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, nous devons engager un travail pour intégrer la fin de vie aux programmes des formations de santé. Le plan prévoira aussi un développement de la prise en charge en ville- vous l'avez souhaité et je partage votre point de vue -, qui sera très vite facilitée par la mise à disposition du Midazolam dès la fin de l'année 2021. Faire connaître la loi pour ne pas avoir un droit bavard et mal appliqué, c'est un impératif, mais ce n'est pas le seul. Il y a également un enjeu de moyens. À cet égard, le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale devra intégrer des mesures nouvelles pour augmenter la dotation socle des soins palliatifs. Ce sera au législateur de définir ces moyens et ce cap. Au chapitre des moyens, je ne peux pas pas ne pas rappeler que le Ségur de la santé a prévu pas moins de 7 millions d'euros pour l'appui sanitaire aux Ehpad, ceux-ci incluant la mise en place d'astreintes de soins palliatifs. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le débat sur la fin de vie est un débat essentiel. Il mérite évidemment de l'apaisement, du sang-froid et tout le temps nécessaire à un sujet de société aussi important. Nous sommes aujourd'hui encore en plein combat contre la crise virale, avec un système de santé totalement mobilisé, au front, et des mesures sanitaires qui pèsent lourdement sur le quotidien de nos concitoyens. Pour le dire autrement, je ne pense pas que le moment choisi pour modifier le régime juridique de la fin de vie soit opportun, mais je sais que nos échanges permettront de nous fixer un horizon et de renforcer les dispositifs existants. L'une des grandes avancées de la loi Claeys-Leonetti est d'avoir permis un accompagnement juste et adapté des personnes en fin de vie. Beaucoup de professionnels des soins palliatifs considèrent d'ailleurs que cette loi, si elle était correctement appliquée, suffirait à protéger l'autonomie de chaque individu face à la mort. Il y a des situations de grande détresse qu'il faut entendre et pour lesquelles nous devons trouver des solutions, dans leur immense majorité déjà mobilisables dans notre droit. Sur un sujet aussi sensible, je le répète, sans porter le moindre jugement sur les demandes, dont le fondement relève de l'intimité la plus profonde, sans dogmatisme aucun,

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la question de la fin de vie « interroge chacune et chacun d'entre nous sur son rapport intime à la vie et à la mort.

résonnent dans notre hémicycle alors que nous examinons cette proposition de loi. La fin de vie est un sujet de société majeur, qui intéresse et mobilise nos concitoyens. En témoignent les dernières enquêtes d'opinion réalisées, selon lesquelles 89 % des Français sont favorables à une évolution de la législation. de la législation. C'est pourquoi je souhaite remercier l'auteure de cette proposition de loi, Marie-Pierre de La Gontrie, et saluer les travaux de l'association ADMD et de son président, Jean-Luc Romero, dont je connais l'engagement. Il est présent aujourd'hui. Car si le droit a connu des évolutions importantes ces dernières années, nous constatons d'importantes disparités sur notre territoire. Nous ne pouvons rester muets face aux difficultés juridiques de mise en oeuvre de notre législation, qui conduit au départ de nombreux Français à l'étranger lorsque leurs ressources le leur permettent, créant des inégalités liées aux ressources de chacun. Pour celles et ceux qui en ont les moyens, être contraint de se rendre à l'étranger signifie bien souvent une fin de vie loin de leur pays, sans la présence de leurs proches et de leur famille, privés d'un accompagnement moral si important. Comme l'indique le CESE dans un avis rendu en 2018, l'offre de soins palliatifs demeure insuffisante dans notre pays et inégalement répartie sur notre territoire, je pense notamment aux outre-mer. Au total, cela a été dit, vingt-six départements, dont Mayotte et La Réunion, ne sont pas dotés d'unités de soins palliatifs. Il convient donc de renforcer cet accès afin de permettre à nos concitoyens d'avoir une fin de vie digne et conforme à leurs souhaits. Mes chers collègues, comme nos concitoyens, nous avons tous été confrontés à la perte d'un proche. Nous connaissons le sentiment d'impuissance que l'on éprouve durant ses derniers instants, auquel s'ajoute une profonde tristesse. Que dire alors, Que dire alors, et je reprends les mots de Jean-Luc Romero, lorsque ce proche vit ses derniers instants dans la souffrance, sans avoir pu choisir « le moment et la manière d'éteindre soi-même sa propre lumière » ? Pour lui, pour nous, nous ne pouvons évidemment pas l'accepter. Il s'agit là d'un grand chantier que nous devrons conduire dans les mois et les années à venir, et je sais la mobilisation sur cette question de la majorité présidentielle et du Gouvernement, notamment par la voix du garde des sceaux, et, plus largement, sur l'ensemble des bancs de nos assemblées. À cet égard, et comme le soulève l'ensemble des acteurs, le renforcement d'unités mobiles de soins palliatifs constituerait une première piste de réflexion. Cette proposition de loi, qui prévoit d'inscrire dans le code de la santé publique le droit à l'aide active à mourir dans les cas de pathologies au caractère grave et incurable avéré et infligeant une souffrance physique ou psychique, constitue une réponse aux difficultés que pose notre législation. Elle pose également le sujet essentiel des directives anticipées, en permettant leur développement et en instaurant un fichier national les recensant, ce qui constitue une avancée non négligeable que nous tenons à saluer et à soutenir.

à la conception que nous nous faisons de la vie et de la mort. C'est pourquoi chaque membre du groupe RDPI votera ce texte en son âme et conscience. À titre personnel, comme l'écrasante majorité de mon groupe, je voterai pour. La parole est

exceptionnellement, je débuterai par ce qui devrait être la fin de mon intervention : le groupe du RDSE est partagé sur cette proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité. partagé, car ce texte, au-delà des schémas partisans classiques, touche à ce que nous avons de plus intime, notre rapport à la mort. Il fait rejaillir des situations que nous avons pu connaître pour nos parents, nos amis ou nos proches et qui restent parfois douloureuses. partagé aussi, car une « bonne mort », pour reprendre l'étymologie du mot euthanasie, ne se décrète pas. Nous pouvons chacun avoir une interprétation de ce qu'elle peut être ou non et cette conception peut évoluer tout au long de notre vie. À cet égard, je tiens à saluer à mon tour la mémoire de Paulette Guinchard-Kunstler, ancienne secrétaire d'État socialiste, décédée après avoir eu recours à un suicide assisté en Suisse, alors même qu'elle s'était opposée à cette pratique en 2005. Son choix de faire connaître sa décision est une preuve de courage sans commune mesure et force le respect.

Car au-delà de l'affirmation des droits existants, il nous faut les garantir pleinement, et force est de constater que ce n'est pas le cas. Concernant les soins palliatifs d'abord, si des progrès ont récemment été effectués, l'on estime que près de 20 % des personnes qui pourraient les solliciter n'y ont pas accès. Les raisons en sont nombreuses : l'absence d'information sur ces soins, le manque de formation des personnels de santé, mais aussi une grande disparité territoriale, selon que l'on réside dans une métropole ou dans un territoire rural- j'en suis témoin. Ce constat est partagé par le Conseil économique, social et environnemental qui, dans son rapport de 2018 intitulé, indiquait que l'offre de soins palliatifs est « insuffisante et inégalement répartie ». C'est d'autant plus vrai qu'un nombre croissant de Français fait le choix du maintien à domicile. Ce que j'évoque concernant les soins palliatifs est également valable pour les directives anticipées. Créées en 2016, elles devaient permettre de connaître les volontés en termes de soins médicaux d'une personne devenue inconsciente ou incapable de s'exprimer. L'objectif était d'éviter les drames familiaux, comme dans l'affaire Vincent Lambert, dont les proches se sont déchirés durant des années au sujet du consentement qu'aurait ou non donné celui-ci. À cet égard, on peut regretter que des affaires comme celle-ci n'aient pas incité les pouvoirs publics à lancer une vaste campagne d'information au sujet des directives anticipées. Au fond, c'est l'absence d'effectivité de la loi actuelle qui fait que certains d'entre nous s'interrogent sur l'opportunité de franchir l'étape supplémentaire qu'est l'ouverture du droit de mourir dans la dignité. D'autres de nos collègues sont convaincus qu'il faut passer à cette étape d'abord parce qu'ils sont attachés à la liberté individuelle et pensent que, lorsque les circonstances le justifient, chacun doit pouvoir choisir sa mort ; ensuite parce qu'ils estiment que la sédation profonde et continue, tout comme la notion de non-acharnement thérapeutique, qui consiste au final à endormir et à laisser mourir par l'arrêt des traitements, ne permet pas de garantir une fin de vie digne aujourd'hui ; enfin parce qu'ils considèrent que le cadre juridique posé par l'article 2 est suffisamment rigoureux, ce que l'on ne peut nier. En prévoyant que le patient doit être en phase terminale ou avancée d'une affection pathologique ou accidentelle, que celle-ci doit être incurable, le législateur apporte de véritables garanties aux plus sceptiques d'entre nous. Il le fait encore lorsqu'il prévoit que pour bénéficier de ce droit, cette affection doit infliger une souffrance physique ou psychique inapaisable, insupportable ou plaçant le malade dans un état de dépendance qu'il estime incompatible avec sa dignité. Enfin, ces garanties sont données lorsque les médecins doivent consulter leurs confrères et émettre un avis collégial sur la mise en oeuvre de l'aide active à mourir. Nous défendrons d'ailleurs un amendement visant à renforcer cette collégialité. Comme je vous l'ai dit au début de mon propos, le groupe du RDSE reste partagé sur cette proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le philosophe Sully Prudhomme disait : « Il est bon d'apprendre à mourir par volonté, non d'un coup traître. [ ...] Qui sait mourir n'a plus de maître. La covid-19 a malheureusement été le maître de nombreuses décisions concernant la fin de vie ces derniers mois. Or, en ce domaine, comme en beaucoup d'autres, les inégalités territoriales sont fortes et il n'est pas excessif d'avancer qu'on meurt, encore trop souvent, dans de mauvaises conditions en France. La pandémie fut en quelque sorte un miroir grossissant de toutes ces difficultés et des souffrances qu'elles engendrent. Elle a accentué les problèmes de pénurie de médicaments, notamment de Midazolam, utilisé pour les sédations terminales. Les personnes en fin de vie n'ont pas eu accès à ce médicament, conservé pour la réanimation, et un traitement de substitution, le Rivotril, leur a été administré dans les Ehpad. son utilisation, dans le cadre de l'urgence sanitaire, n'a malheureusement pas étendu son emploi à domicile. Enfin, pendant de très longues semaines, les visites des proches et des familles ont été interdites pour les personnes en fin de vie, entravant voire empêchant un accompagnement et une présence indispensables. Cette proposition de loi en faveur de la légalisation de l'euthanasie, du suicide assisté et d'un accès universel aux soins palliatifs est plus que jamais d'actualité. Même si la loi dite Claeys-Leonetti constitue une avancée avec l'instauration du droit à la sédation profonde et continue, elle est insuffisante et mal connue, tant par les patients que par les soignants. Les auditions organisées par Michelle Meunier ont par ailleurs confirmé que les directives anticipées étaient rares. Le Conseil économique, social et environnemental avait fait état en 2018 des difficultés de mise en oeuvre du droit à la sédation profonde. Celles-ci ne sont toujours pas résolues et persistent, en raison notamment de problèmes d'ordre médical, juridique et éthique. Actuellement, l'état du droit conduit de nombreuses personnes à partir à l'étranger, quand elles en ont les moyens, pour y terminer leur vie conformément à leurs souhaits. Cette discrimination par l'argent est intolérable ! Nous ne pouvons que regretter en la matière l'absence de position commune en Europe, où les législations connaissent de profondes disparités en matière d'euthanasie active. Faut-il redire que cette proposition de loi répond à une demande forte des Français, qui souhaitent que la législation évolue afin d'autoriser les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie des personnes qui en font la demande ? Elle constitue un progrès.

pour tout acte médical, une clause de conscience. Pour notre groupe, la meilleure prise en considération des volontés des patients et un plus grand respect des conditions de fin de vie sont des éléments fondamentaux pour garantir la liberté et l'égalité des droits devant la mort. D'ailleurs, le texte que nous examinons reprend les termes d'une proposition de loi déposée en 2011 par le groupe communiste, sous l'impulsion de Guy Fischer et Annie David, alors présidente de la commission des affaires sociales. Parallèlement, comment ne pas s'interroger sur le développement des soins palliatifs, qui a hélas ! pris beaucoup de retard, puisque, entre 2015 et 2018, seuls 210 lits en unités de soins palliatifs ont été créés, ainsi que 6 équipes mobiles. Le 13 février dernier, l'IGAS a publié un rapport très critique sur l'état des soins palliatifs. Résultat, l'offre « est globalement insuffisante », de fortes disparités régionales étant constatées, « et ne répond pas bien à la demande de la population qui devrait recevoir des soins palliatifs Pour améliorer la fin de vie et mettre en oeuvre un droit à mourir dans la dignité, il faut donc faire évoluer la loi, mais également renforcer le développement des soins palliatifs, recruter des professionnels spécialisés, donc bien formés. J'ai bien entendu votre engagement,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je tiens à remercier notre rapporteure pour la qualité des travaux qu'elle a menés. Comme beaucoup des orateurs qui sont intervenus et qui s'exprimeront aujourd'hui dans le cadre de cette discussion générale, c'est avec beaucoup de modestie que je prendrai la parole au nom de mon groupe sur un texte qui, par essence, ne peut pas faire l'objet d'une position commune. Dès lors, le vote du groupe Union Centriste sur l'ensemble de cette proposition de loi sera nécessairement partagé. Toutefois, une chose nous rassemble et nous indigne à la fois, et je ne crois pas m'avancer si je dis que cela nous rassemble tous ce matin. En effet, et pardonnez-moi l'expression, « nous mourrons mal en France Un chiffre est particulièrement édifiant, nous sommes plusieurs à l'avoir souligné : vingt-six départements ne disposent pas d'unité de soins palliatifs. Lorsque le décès advient en milieu hospitalier, et en dépit des efforts des personnels, force est de constater que l'environnement du décès ne garantit pas le respect qui est dû à l'intéressé, ainsi qu'aux proches qui l'accompagnent et qui souffrent. Aussi, les membres du groupe Union Centriste profitent de cette tribune offerte par les auteurs de cette proposition de loi pour attirer solennellement l'attention du Gouvernement sur la nécessité de soutenir le maintien et le développement des unités de soins palliatifs,

Cette exigence, monsieur le ministre, permettra d'acculturer les Français aux dispositions toujours trop méconnues de notre droit : nous pensons à la loi du 22 avril 2005, ainsi qu'à la loi du 2 février 2016. Nous estimons qu'un meilleur usage de nos droits, l'élaboration de directives anticipées ou la désignation d'une personne de confiance sont susceptibles d'éviter aux familles des discussions délicates et parfois sources de tensions insoutenables. D'ailleurs, monsieur le ministre, pourquoi ne pas envisager de rendre obligatoire la rédaction de directives anticipées dès l'âge de 18 ans et leur renouvellement tous les dix ans au minimum ? L'usage des nouveaux outils, je pense au dossier médical partagé (DMP) par exemple, devrait permettre d'envisager une telle mesure. Par ailleurs, j'ai été sensible aux propos qu'a tenus en commission la semaine dernière notre collègue Véronique Guillotin. Elle nous a fait part de son expérience de médecin en soins palliatifs à proximité de la frontière belge

Cela confirme assurément nos deux premières exigences : une meilleure connaissance et diffusion de notre droit et la mise en place d'environnements respectueux des familles.

le droit à mourir dans la dignité et, j'ajouterai, dans la sérénité. Aussi, je voterai contre cette proposition de loi qui, par ailleurs, me semble apporter des solutions à un certain nombre de problèmes bien réels, tout à fait délicats, et que l'on ne peut examiner qu'avec les précautions et la finesse auxquelles nous oblige ce sujet.

ce texte ne se situe pas dans le prolongement des lois que j'ai rappelées précédemment. Il prévoit un changement de paradigme en ouvrant la possibilité de recourir au suicide assisté et à l'euthanasie. Je vous rappelle que le législateur a jusqu'à présent toujours fait l'économie de telles dispositions. Il a choisi d'interdire l'acharnement thérapeutique et préféré à l'euthanasie l'usage de médicaments pour soulager les douleurs, bien qu'ils puissent entraîner la mort, ou encore encore d'une sédation profonde en cas de douleur réfractaire aux traitements. Ainsi, nos prédécesseurs n'ont jamais souhaité franchir la ligne qui consisterait à légaliser un acte positif ayant pour seule finalité de tuer une personne ou de lui de se suicider, quand bien même celle-ci serait atteinte d'une maladie grave, incurable et qu'elle en ferait la demande. D'ailleurs, la proposition de loi met en place une fiction juridique, puisque la personne ainsi décédée verrait son décès enregistré comme mort naturelle. Enfin, je m'arrêterai sur l'article 7, qui précise l'ordre de primauté pour déterminer les conditions d'application du dispositif lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, en l'absence de directives anticipées ou de désignation de personne de confiance. La proposition de loi prévoit que sera d'abord consulté le partenaire de vie, sans préciser la durée minimale de la relation. Le partenaire ayant vécu trois mois avec le patient serait donc prioritaire sur l'enfant majeur, mais l'enfant mineur, deux mois avant sa majorité, ne serait pas prioritaire sur ses grands-parents ou ses cousins. Bref, en l'état, cet article ne me semble ni souhaitable ni abouti. Il est surtout susceptible de créer un grand nombre de contentieux, alors que nous recherchons en la matière l'apaisement et la dignité. Malgré ces remarques, je remercie les auteurs de cette proposition de loi, qui nous permettent de débattre d'un sujet important pour notre société, essentiel pour chacun d'entre nous, et d'une importance considérable pour celles et ceux dont les demandes ne trouvent pas encore satisfaction.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le sommet de l'abject se rapproche de jour en jour durant ce quinquennat puisque le Gouvernement a décidé d'abandonner nos anciens en reportant aux calendes grecques le projet de loi Autonomie et grand âge et que les sénateurs socialistes, jamais en retard d'une ignominie, proposent comme alternative à la souffrance en fin de vie l'euthanasie Ce sont les mêmes qui ont aboli la peine de mort pour les assassins qui souhaitent la rétablir pour les innocents dont le seul crime est d'être malades. Depuis un an que nous sommes entrés en crise épidémique, nous avons accepté, de gré, et surtout de force, de mettre à l'arrêt, ou presque, tout un pays pour protéger la vie humaine, dont le prix est inestimable, notamment celle des personnes les plus fragiles, et ce quitte à imposer de grandes souffrances économiques et sociales à toute une nation solidaire. Mais ici, dans ce texte, vous venez balayer tous ces sacrifices en offrant comme perspective macabre aux personnes souffrantes le suicide et donc la mort. Projet nauséabond de matérialistes, plus connus sous le vocable antinomique de « progressistes » ... C'est un mot que vous ne connaissez pas ! ... qui souhaitent éliminer tout ce qui n'est pas utile à la société matérialiste déshumanisée.

Car il y a dans nos établissements de soins palliatifs une médecine tournée vers l'humain dans ses particularités sociales, familiales, physiques et même spirituelles. C'est cette médecine qu'il nous faut soutenir et développer. La souffrance peut faire peur, la volonté de liberté sans frein peut séduire, l'acharnement thérapeutique peut susciter des jamais la mort précipitée ne doit être considérée comme une solution. Les patients ne souhaitent pas mourir, ils souhaitent ne pas souffrir. Alors il faut leur assurer une fin de vie la plus « confortable » possible, c'est l'honneur de notre société ; il y va de notre conscience individuelle, qui ne saurait céder à l'inconscience collective. Vous nous parlez de « suicide assisté », en même temps que nombreux, trop nombreux sont nos compatriotes, notamment paysans, commerçants et représentants des forces de l'ordre, qui se suicident pour fuir la détresse de l'abandon. Il faut une grande ambition de solidarité nationale pour endiguer le phénomène plutôt que de le légaliser. La médecine s'est évertuée jusqu'à nos jours à augmenter l'espérance de vie, faisant de la protection de la vie humaine sa vocation. Vous voulez faire table rase de ce passé en imposant la désespérance de vie, au nom d'une nouvelle liberté. Liberté, voilà un nouveau crime que certains s'apprêtent à commettre en ton nom ! Est-ce cela votre conception d'une société avancée, d'une société moderne, d'une société éclairée ? Tant de Tant de lumière finit par vous aveugler, mes chers collègues, au point de ne plus voir que la vie doit rester au-dessus de tout. Je vous appelle donc, mes chers collègues, à rejeter les arguments fallacieux des tenants de ce texte mortifère. Face à l'offensive des marchands de mort, menée par ces fanatiques de l'IVG et de la mise à mort des malades, le Sénat doit plus que jamais justifier son nom et sa qualité de Chambre haute en étant le rempart infranchissable qui, et quoi qu'il en coûte, protégera toujours la vie

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, comme tout médecin généraliste, j'ai été confronté à la fin de vie de patients atteints de pathologies insupportables ou parfois usés par la vie, désireux d'en finir et l'exprimant régulièrement. Et pourtant ! Je me souviens de Jeanne, me répétant à chaque visite : « Docteur, je veux en finir, je souffre le martyre. » Voulant m'assurer de sa certitude, je lui dis avec compassion que j'étais prêt à répondre à sa volonté. Alors, j'ai vu dans son regard non pas une lueur d'espoir que ses souffrances soient abrégées, mais une crainte de ne plus vivre. Elle m'a demandé timidement, humblement, de reporter à plus tard cette décision lourde. Au fond d'elle-même, elle n'était pas prête. Oui, le doute est permis, la volonté d'un jour n'est pas celle de toujours. Ce dialogue singulier entre un patient et son médecin, s'il doit être encadré par la loi, reste heureusement plus relationnel que législatif. Une loi pour celles ou ceux qui vont mourir, nous l'avons, c'est la loi Leonetti-Claeys » : c'est ce que disait Alain Milon, alors président de notre commission des affaires sociales, au moment de son adoption au Sénat, qui est excusé aujourd'hui. Michel Amiel, corapporteur du texte, citait lui Albert Camus, qui a décrit la mort heureuse, « la tête dans les étoiles ». Dans les faits, ce n'est, hélas ! pas ainsi que les choses se passent, disait-il. Cette proposition de loi s'adresse, elle, à celles ou ceux qui veulent mourir. L'approche éthique est différente, plus sociétale que médicale. Apportera-t-elle l'humanité indispensable à celui qui veut mourir et la sérénité à son entourage et au personnel soignant ? Intimement, je ne suis pas sûr que ce texte réponde à toutes les questions soulevées. Les patients désireux de mourir le veulent-ils vraiment ? Leur volonté est-elle définitive ? N'est-elle pas orientée ? Considérer que l'euthanasie conduit à une mort naturelle, à déclarer comme telle sur le certificat de décès, n'est-ce pas une source de dérive ? Jusqu'où aller dans le respect de la dignité humaine, tellement différente d'un individu à l'autre dans la vie courante, et donc lors de l'inéluctable fin de vie de chacun ? la clause de conscience, n'est-ce pas reconnaître implicitement ne pas savoir jusqu'où aller dans l'aide active à mourir ? Voici quelques propos émanant d'un collectif de médecins en soins palliatifs et de gériatres qui alertent sur ces risques de dérive, vous les avez sûrement lus. Dans les pays où l'aide à mourir est proposée, la critique de l'acte devient difficile, voire impossible. Le respect de la conscience et des volontés des médecins et des malades est mis à mal. Les patients peuvent ressentir une pression sociale, parfois même familiale, les poussant à demander une mort anticipée. Sommes-nous dès lors toujours dans la thématique du choix ?

Évaluons d'abord son application. Nous verrons vite qu'elle n'est pas suffisamment mise en oeuvre, parce que pas encore assimilée, et pour cause ! Il y a très peu de directives anticipées ; M. le ministre l'a loi préconisait un développement des services de soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, ce qui n'a toujours pas été fait. Cela fait partie de ces innombrables inégalités territoriales, qui vont de la naissance au dernier jour, et dont tout le monde parle,

avec l'augmentation progressive de l'espérance de vie et l'évolution de notre société, les questions d'euthanasie agitent et animent régulièrement nos débats sociétaux, ainsi que nos bonnes consciences. En 2005, la loi Leonetti a permis de faire un grand bond en avant en autorisant toute personne en phase terminale d'une maladie incurable à décider de limiter ou de stopper ses traitements.

Rappelons que ce sont des soins actifs et positifs, avec administration d'antalgiques, de corticoïdes ou poursuite de certains traitements, mais dans le seul objectif de soulager le patient jusqu'à la fin. Il n'est aucunement question de provoquer le décès par injection d'une substance létale. L'usage de certains antalgiques, notamment de la famille des opiacés, à forte dose, est autorisé pour des raisons d'efficacité, même s'ils peuvent accidentellement entraîner le décès prématuré du patient. Il s'agit donc de préserver la dignité de la personne en lui épargnant autant que faire se peut douleurs et souffrances psychologiques. En 2016, un nouveau pas a été franchi avec la loi Claeys-Leonetti, qui a introduit les notions fondamentales de « directives anticipées » et de « sédation profonde et continue ». Après accord du patient et de la famille, le médecin, à l'aide de produits anesthésiques, peut altérer la conscience du patient arrêter les traitements, afin d'entraîner un décès en douceur. La différence fondamentale avec le suicide assisté est simple : ce dispositif s'adresse non pas à des personnes qui veulent mourir, mais à des personnes qui vont mourir. La loi Claeys-Leonetti a marqué un progrès fondamental dans le traitement des maladies incurables. Il convient désormais- vous l'avez rappelé fort justement, monsieur le ministre -de la faire connaître, de la relayer sur le terrain et de veiller à son application. Un nombre trop important de médecins et de soignants refusent encore, sous prétexte de craintes souvent injustifiées, de mettre en oeuvre ses dispositions. Cette loi a gravé dans le marbre des actes que les médecins pratiquaient déjà dans l'intérêt du patient et des familles, avec beaucoup de compassion et d'humanisme. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui nous invite, avec le suicide assisté, à un changement de paradigme fondamental. Il ne s'agit pas simplement, comme certains le pensent, de déterminer si nous y sommes prêts il s'agit de savoir si nous considérons qu'une telle option constitue, ou non, un choix de société souhaitable. Un tel débat ne peut pas se résumer en dix articles. Un encadrement juridique bien plus détaillé

Très beau sujet de réflexion pour les juristes et les assureurs ! Mes chers collègues, à mon sens, cette proposition de loi ne permet pas d'évaluer et d'encadrer correctement tous les cas de souffrances psychologiques ou physiques qui relèveraient d'un suicide assisté. Chaque cas est unique et devrait être traité individuellement, après avis d'un comité d'éthique médicale. Les équipes de soignants le savent : judicieusement appliquée et adaptée en fonction de certaines circonstances, permet de traiter la grande majorité des cas. Elle me paraît largement suffisante et satisfaisante pour l'heure. Laissons faire les médecins. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants - République et

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question du droit individuel à bénéficier de l'aide active à mourir, dans un cadre strictement défini et contrôlé, s'invite régulièrement dans l'actualité.

Il nous faut donc comprendre ce qui insiste comme ce qui résiste dans ce débat en France. L'objection première est qu'un tel choix résulterait d'un défaut d'accompagnement de qualité de la fin de vie, d'une non-application ou d'une mauvaise application des lois existantes, de l'absence d'unités de soins palliatifs. Certes, on meurt mal en France. Et, effectivement, les soins palliatifs attendent depuis trois ans un nouveau plan. Les fermetures, toujours en cours, de dizaines de milliers de lits de spécialités médicales, en cancérologie, en pneumologie, en gériatrie, où l'accompagnement de type palliatif s'exerçait, ont diminué l'offre de lits palliatifs.

D'ailleurs, cette proposition de loi réaffirme le droit effectif universel à accéder à des soins palliatifs dans tous les départements, proportionnellement à leur population.

ni sa conception personnelle d'une mort digne. Ce qui insiste donc, c'est la demande que la société entende et respecte le choix, irréductible à l'individu, de décider du moment de partir, et qu'elle permette l'effectivité de ce choix individuel dans le cadre collectif qu'elle a défini. À l'inverse,

Ce refus condamne souvent à des suicides violents et prématurés, à des pratiques illégales à la seule discrétion des médecins- faut-il dire « du pouvoir médical » ? -, au départ à l'étranger ou à des fins de vie vécues comme indignes par la personne et son entourage. Ce que le législateur reconnaît par cette proposition de loi, quand la médecine elle-même se retire, c'est le droit de chacun à être aidé pour choisir- j'emprunte cette expression -le moment d'« éteindre la lumière ». Paulette Guinchard-Kunstler a souhaité que son suicide assisté soit connu dans l'espoir de faire bouger les lignes. Rappelons que, après la première loi Leonetti, défenseuse du développement des soins palliatifs,

Je pense que tout le monde a droit à ce cheminement de liberté et je vous invite à voter la loi le permettant. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question de la fin de vie anime régulièrement le débat public, ravivée à chaque exemple douloureux d'une fin de vie de souffrances pour un patient et sa famille. Ces débats ont permis des avancées législatives significatives en matière d'accompagnement pour une fin de vie digne, en particulier grâce aux lois Leonetti et Claeys-Leonetti, votées respectivement en 2005 en 2005 et en 2016. Mais pour les malades et leurs familles, pour les associations qui les soutiennent et pour un grand nombre de nos concitoyens, le dispositif législatif actuel demeure insuffisant. Bien sûr, des mesures telles que l'interdiction de l'obstination déraisonnable, la désignation d'une personne de confiance ou encore l'instauration des directives anticipées constituent des avancées concrètes, quoique parfois méconnues par nos compatriotes, qui y ont encore peu recours. La législation existante se borne en outre à limiter le choix des patients entre une sédation profonde et continue, souvent suivie d'une lente agonie, et un thérapeutique entraînant trop fréquemment des souffrances insupportables. La proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, que je suis heureux d'avoir cosignée, prend ainsi tout son sens. Elle s'inscrit dans un contexte où la demande des Français d'obtenir le droit de mourir dans la dignité est unanime. Comme cela a été rappelé, selon un sondage de l'institut Ipsos de mars 2019, 96 % des personnes interrogées sont favorables à la reconnaissance d'un droit à l'euthanasie. Un tel pourcentage est éloquent et ne peut pas nous laisser indifférents Cette proposition de loi vise en outre à rompre avec un système aujourd'hui inégalitaire face à la fin de vie, car seules les personnes qui en ont les moyens peuvent décider de partir à l'étranger afin d'y terminer leur existence conformément à leurs souhaits. Soulignons à cet égard que, après les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, un quatrième pays européen, le Portugal, vient d'adopter, le 29 janvier dernier, une loi dépénalisant l'euthanasie.

Si comparaison n'est pas raison, nous ne pouvons pas faire fi de cette évolution sociétale, qui s'étend désormais de part et d'autre de nos frontières. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise ainsi à mettre en place un dispositif juste et sécurisant pour les malades et les praticiens en ouvrant enfin le droit pour les patients de solliciter l'aide active à mourir, dans un cadre législatif rigoureux. texte reconnaît à tous les citoyens le droit de pouvoir choisir de mourir dans des conditions dignes et strictement conformes à leurs souhaits. Mes chers collègues, l'heure de la mort fait légitimement appel pour chacun d'entre nous à des sentiments profonds et personnels, à des convictions intimes. C'est pourquoi il n'est jamais aisé de légiférer en la matière. Pourtant, et comme d'autres l'ont fait avant nous au sein de la Haute Assemblée, nous pouvons choisir de donner à chacun de nos compatriotes le droit de maîtriser les conditions de sa mort, comme chaque être humain est en droit de choisir les modalités de sa propre vie. Ce texte prévoit donc d'inscrire dans le code de la santé publique le droit de bénéficier de l'aide active à mourir. Il en définit précisément les conditions de mise en oeuvre, ainsi que les critères permettant aux patients de pouvoir y avoir recours. Considérant qu'il ne peut pas y avoir de fin de vie digne sans qu'un environnement adapté et suffisant soit mis en place autour du patient et de sa famille, la proposition de loi détermine également les modalités de désignation des personnes de confiance et renforce la prise en compte des directives anticipées, en réaffirmant leur caractère contraignant pour l'équipe soignante et en actant la création d'un registre national automatisé. Elle permet par ailleurs à la personne de confiance de demander l'aide active à mourir lorsque le patient a indiqué vouloir en bénéficier dans ses directives anticipées et alors qu'il se trouve hors d'état d'exprimer sa volonté. Enfin, il ne saurait y avoir d'ouverture de droits nouveaux en matière de fin de vie sans que l'on offre à nos concitoyens la garantie pour tous, où qu'ils se trouvent sur le territoire national et dès lors que leur état de santé le requiert, d'un accès effectif aux soins palliatifs. Cette proposition de loi institue donc un droit universel d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement, dont la mise en oeuvre devra faire l'objet d'un rapport annuel de la part du Gouvernement. Les inégalités territoriales restent en effet criantes en la matière et nécessitent des moyens financiers et humains à la hauteur des enjeux. Mes chers collègues, au-delà de nos conceptions philosophiques et de nos appréciations personnelles et intimes, de notre propre rapport à la mort, le texte soumis aujourd'hui à notre examen constitue fondamentalement une loi de liberté. Il n'impose rien, mais il vise à permettre à chacune et chacun d'avoir la faculté ultime de choisir sa fin de vie. C'est la raison pour laquelle, au-delà de nos sensibilités politiques,

Aujourd'hui, nous examinons une proposition de loi instaurant un droit à mourir, et cette pensée antique s'inscrit parfaitement dans le débat actuel. En effet, ce texte a été présenté afin d'offrir aux patients volontaires une mort digne, grâce à l'euthanasie ou au suicide assisté. Lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales, la présidente Catherine Deroche soulignait que la dignité d'un homme était préservée jusqu'à son dernier souffle, malgré la déchéance physique, que nous ne pouvons pas considérer comme indigne. La question suivante se pose : l'accélération de la fin de vie est-elle un moyen de préserver la dignité humaine ? Mon âme de médecin me fait penser que non. L'article 2 de la proposition de loi édicte un certain nombre de critères qui permettent aux médecins d'apprécier la recevabilité de la demande d'aide active à mourir. Celle-ci renvoie à la notion de « dernière volonté ». Or comment s'assurer que ce souhait constitue une volonté définitive ? Toute erreur de jugement de la part d'un patient souhaitant bénéficier d'une aide active à mourir serait irréversible. À cet égard, l'exemple évoqué par René-Paul Savary est édifiant. En dépit de la clause de conscience proposée, le médecin engagerait sa responsabilité morale en acceptant ou en refusant un tel acte. La loi est-elle en mesure d'apporter des réponses appropriées à toutes les situations ? diffère selon les contextes de vie et d'hospitalisation. Il me paraît audacieux de généraliser une pratique aussi exceptionnelle qu'intime. Par ailleurs, l'article 4 de la proposition de loi définit le régime de la personne dite de confiance, en prévoyant un classement « par ordre de préférence Mes chers collègues, je suis père de quatre enfants. Je vous assure être dans l'incapacité la plus totale d'établir un ordre de préférence entre eux. La position que je défends aujourd'hui semble être similaire à celle du Comité consultatif national d'éthique, qui rappelait en 2019 que la loi n'avait pas vocation à arbitrer ou à résoudre les questions éthiques « nécessairement déchirantes » liées à la fin de vie, mais qu'elle devait poser « un cadre nécessaire pour la cohésion et la solidarité entre les individus dans une société En revanche, je salue l'apport de l'article 9 de la proposition de loi, qui instaure un droit universel aux soins palliatifs. Ce texte nous accorde ainsi la possibilité de dresser un bilan de l'offre de soins palliatifs en France, qui reste bien trop insuffisante à ce jour. Je partage pleinement l'objectif de rendre effectif le droit de bénéficier de ce type de soins. Il me paraît essentiel d'augmenter les moyens afin de permettre au système hospitalier d'accueillir davantage de patients en fin de vie. Ce mardi, Jean Castex a annoncé la mise en oeuvre du deuxième volet du Ségur de la santé, à savoir le « lancement d'une nouvelle politique d'investissements dans le système de santé ». Ce plan est composé d'une enveloppe de 19 milliards d'euros, mais les soins palliatifs n'y sont pas mentionnés. Monsieur le ministre,

une proportion encore très faible, cinq ans après l'adoption de la loi Claeys-Leonetti. Par ailleurs, 54 % des personnes interrogées ne souhaitent pas en rédiger. Ces chiffres nous invitent à tirer la conclusion selon laquelle la majorité des Français ne semblent pas attendre une évolution législative dans ce domaine. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous voterons contre cette proposition de loi. Enfin, comme je pense que ce sont nos expériences personnelles ou professionnelles qui forgent notre conviction intime sur le sujet, des miennes. Voilà quelques mois, pour la première fois dans ma carrière professionnelle, j'ai annoncé à une jeune patiente qu'elle allait mourir. Elle m'a demandé le droit à vivre dans la dignité.

Nous constatons tous, me semble-t-il, que trop de personnes dans notre pays meurent insuffisamment soulagées, insuffisamment apaisées et, pour tout dire, insuffisamment respectées dans leurs derniers instants.

Ce sera la responsabilité du Gouvernement et la nôtre en tant que parlementaires. Certains estiment qu'une bonne application de notre législation actuelle suffirait à résoudre de telles situations.

pour lesquels la législation actuelle n'est pas adaptée. Ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais ils le sont suffisamment pour que le législateur remette le sujet à l'ordre du jour et fasse évoluer la loi.

Il est difficile d'expliquer à des familles dont un membre souffre que le seul horizon proposé se résume à une lourde thérapie n'ayant pour fonction que de faire gagner quelques jours de vie supplémentaires. Car de quelle vie parle-t-on ? Une vie faite de souffrances, de douleurs, d'espoirs déçus ! Le besoin impérieux de soulager ceux qui souffrent et ceux qui les accompagnent nous oblige à légiférer. Le droit à mourir dans la dignité et à bénéficier d'une fin de vie apaisée est attendu par une immense majorité de nos concitoyens. En effet, en 2014, un sondage réalisé par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité révélait que 96 % des Français étaient favorables à l'euthanasie.

Jean-Yves Goffi, professeur de philosophie à l'université Pierre-Mendès-France, à Grenoble, spécialiste des questions de bioéthique, explique que l'argument fondamental est le droit ou non de disposer de sa vie. C'est l'argument libéral de la souveraineté sur soi-même. Il est tyrannique de limiter la liberté d'action d'un individu qui, agissant en toute connaissance de cause, ne cause aucun tort aux autres. Or, depuis le début des années 2000, la législation française a déjà connu à plusieurs reprises des évolutions. Pourtant, les Pourtant, les questions liées à la fin de vie n'ont pas toutes trouvé une réponse. La loi Leonetti-Claeys est encore insuffisante. En l'état actuel du droit, de nombreuses personnes en sont réduites à partir à l'étranger, quand elles en ont les moyens, pour y terminer leur vie conformément à leurs souhaits. D'autres parviennent à obtenir d'un médecin une assistance active à mourir. Cela conduit à des inégalités considérables face à la fin de vie. Mes chers collègues, cette proposition de loi répond à la nécessité de faire évoluer la législation vers une aide active à mourir. C'est la seule voie qui permette d'ouvrir et de faciliter le libre choix de nos concitoyens. La parole est à Mme

cette proposition de loi pour relayer le témoignage d'une famille. Mme Colette Delcourt, habitant le Pas-de-Calais, avec qui j'ai échangé, a vécu une expérience qui doit nous conduire à nous interroger sur les conditions actuelles de fin de vie et, plus précisément, sur la fin de vie des personnes en situation de handicap mental. La loi Leonetti ne prévoit rien concernant le consentement des personnes handicapées mentales. pas la douleur infinie que peut représenter pour une mère le fait d'accepter d'être à l'origine de la fin de vie de son fils. Mme Delcourt a cherché des réponses et des accompagnements,

de loi. Comment est-il possible d'adapter le recueil du consentement des personnes handicapées mentales ? Vers qui orienter les familles pour les accompagner et les conseiller ?

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi devrait être la locomotive des grands changements de notre société,

L'euthanasie et le suicide assisté sont des dispositifs législatifs déjà en place dans certains pays d'Europe, comme mes collègues l'ont déjà indiqué. Disons-le, en la matière, la France a encore du retard par rapport à ses voisins. Deux textes, la loi Leonetti de 2005 et la loi Claeys-Leonetti de 2016, prévoient des dispositions à ce sujet, mais ils ne font que préciser les modalités d'accompagnement médical de la fin de vie, en se fondant sur deux piliers : la lutte conte l'acharnement thérapeutique et l'amélioration des conditions de vie du patient en fin de vie. Très concrètement, ces textes ne garantissent en aucun cas la possibilité pour une personne

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la semaine dernière, Paulette Guinchard-Kunstler nous a quittés à l'âge de 71 ans, en nous adressant un dernier message. La première fois que l'on croisait Paulette, on était enveloppé par sa gentillesse, sa bonté, sa bienveillance, sa gouaille, son regard franc et rieur que ne venaient pas troubler les longues mèches grises qui lui couvraient la moitié du visage. Fille de paysan, issue d'une fratrie de huit enfants, elle s'engage dans sa ville professionnelle comme infirmière en psychiatrie auprès d'enfants autistes. Elle s'engage aussi en politique, dès ses 20 ans, d'abord par la voie du syndicalisme agricole catholique, puis au PSU de Michel Rocard et, enfin, au PS de François Mitterrand, auquel elle restera fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Maire, députée, secrétaire d'État, auteure de la grande loi sur l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), Paulette Guinchard-Kunstler était malade depuis près de quinze ans. Elle savait, par son expérience familiale, à quoi la conduirait cette maladie dégénérative incurable. Je m'en étais entretenu avec elle alors que j'étais encore ministre. À cette femme qui a tant souffert et tant fait pour son pays, qu'avons-nous répondu ? Rien. Va mourir en Suisse. Ici, ton corps ne t'appartient pas Ce scandale que constitue la situation d'abandon d'une immense majorité des personnes en fin de vie dans des conditions insupportables nous concerne tous, mes chers collègues. Le temps s'écoule sans faire de bruit. La décision de Paulette Guinchard-Kunstler doit nous conduire à voter cet article 1. voter cet article 1. Nous permettrions ainsi à chacun de vivre avec un sentiment de dignité jusqu'à la fin de ses jours. Nous parlons d'un droit fondamental de la personne humaine, d'une nouvelle liberté : la liberté de choisir. Mes chers collègues, qui sommes-nous pour vouloir entraver « Les grandes peurs périssent d'être reconnues », dit Camus. Et que cette peur-là est grande, je vous le concède ! Commençons par pouvoir décider en conscience des conditions de notre propre fin de vie et méditons

L'aimer, c'était la respecter. L'aimer, c'était la laisser partir. » Mes chers collègues, je voterai en conscience l'article 1de la proposition de loi de Mme de La Gontrie. M. Jean-Claude Tissot, sur l'article. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie représente la conquête d'un droit fondamental la possibilité pour chacun d'entre nous de mourir dans la dignité. Inscrire dans le code de la santé publique le droit à l'aide active à mourir est une mesure d'égalité. En effet, en l'état actuel du droit, de nombreuses personnes sont amenées à partir à l'étranger, quand elles en ont les moyens et la possibilité, pour y terminer leur vie conformément à leurs souhaits. À l'inverse, les personnes qui n'en ont pas les moyens financiers et humains ou celles qui sont dans l'impossibilité de se déplacer doivent faire face aux pires difficultés dans leurs derniers jours. Sur ce sujet, les inégalités sont considérables et elles sont inacceptables pour notre pays. notre pays. Dans son étude sur la révision des lois de bioéthique, le Conseil d'État a lui-même signalé des inégalités territoriales très inquiétantes dans l'accès aux soins palliatifs- n'oublions pas, cela a été dit, que vingt-six départements français n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Il convient également de rappeler que la France se classe parmi les pays d'Europe ayant les taux de suicide les plus élevés chez les personnes âgées. Le « mal vieillir » est une réalité que le législateur doit prendre en compte dans sa globalité. Nous devons permettre le choix égal et encadré entre continuer à vivre, en bénéficiant de soins palliatifs effectifs, et avoir accès au suicide assisté. Les deux ne sont pas opposés et préservent la dignité de chacun. Mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de cet article 1 pour rendre pleinement effectif le droit à mourir dans la dignité.

Il y a deux dangers à éviter : se suicider quand il ne le faut pas et ne pas se suicider quand il le faut ». Et il a dit à ses esclaves, quelque temps avant de se suicider lui-même

Aujourd'hui, le débat est le même. Depuis deux mille ans, notre humanité remue ces questions au plus profond d'elle-même parce qu'elles donnent sens à notre vie. Vous me permettrez d'évoquer ce que mon grand-père m'a enseigné et l'image de ces résistants qui, sous la torture, ont préféré se suicider, se défenestrer, pour échapper au sort indigne qui leur était réservé. Jusqu'à la fin de sa vie, mon grand-père a lui aussi souhaité pouvoir disposer de sa vie et de sa mort. Je tente de conduire mon existence selon mes convictions humanistes. Je veux décider de ma mort et je vous demande de m'en donner le droit au nom de mon humanité, au nom de l'humanité que chacun d'entre nous porte en lui. En choisissant ma mort, je veux transmettre aux générations futures l'exigence de la condition humaine, parce que, ma certitude, c'est que c'est la mort qui donne du sens à la vie. La

Ce n'est plus possible. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour les annonces que vous avez faites tout à l'heure et je serai très vigilante sur les montants qui seront attribués aux soins palliatifs. Je remercie

Vous avez aussi parlé des directives anticipées. Vous avez raison, très peu de Français en ont rédigé,

la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,

J'espère que le Parlement français prendra ses responsabilités et nous soulagera, nous, en Belgique, car j'aimerais que vous voyiez l'état déplorable dans lequel arrivent certains de vos compatriotes qui font des centaines de kilomètres pour être libérés. Ce n'est pas normal Le docteur de Locht vous remercie ; je vous remercie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à mon tour, je remercie Marie-Pierre de La Gontrie de son initiative et, par la même occasion, je salue les associations et les bénévoles qui plaident sans relâche en faveur de l'évolution de la législation vers une aide à mourir.

ajoute une seconde condamnation à celle de la maladie : vivre l'épreuve de leur propre déchéance. Annoncer sa volonté d'en finir, en disant sa douleur, n'est pas un choix facile ; il faut du courage. On le fait pour soi-même et pour ceux qu'on aime. En retour, aimer cette personne, c'est la comprendre et l'accompagner.

l'article IV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui

Je sais bien qu'il existe un certain nombre de lois, nous les avons évoquées : la loi Leonetti de 2005, la loi Claeys-Leonetti de 2016. Pour autant, les fins de vie auxquelles nous assistons sont parfois inhumaines.

avoir l'assurance que, jusqu'au dernier souffle, la dignité que l'on a essayé de construire tout au long de sa vie sera respectée.

C'est la raison pour laquelle je souhaite, mes chers collègues, que nous puissions laisser la possibilité au Gouvernement et à la majorité à l'Assemblée nationale, le moment venu,

La loi Claeys-Leonetti, votée en 2016, a déjà profondément modifié les dispositions applicables en matière d'accompagnement de la fin de vie. Cependant, il est globalement reconnu que cette loi n'est pas encore suffisamment bien appliquée. En conséquence, il semble plus judicieux de s'attacher à la faire appliquer plutôt que de modifier les dispositions déjà applicables, mais non encore appliquées. Je le répète, dans de nombreux cas, cette loi est largement suffisante. J'ajoute que, dans notre pays, qui est en avance par rapport à d'autres où rien n'est prévu,

uniformément appliquée sur le territoire, il n'en demeure pas moins qu'elle comporte des lacunes. Elle n'offre pas de réponse satisfaisante dans certaines situations dans lesquelles les patients ne peuvent pas bénéficier de la sédation profonde et continue jusqu'au décès parce qu'ils ne qu'ils ne remplissent pas les critères, comme l'imminence du décès, par exemple. Dans ces conditions, les patients sont contraints soit de se rendre à l'étranger, soit de se résigner à une dégradation inéluctable et gravement incapacitante de leur état de santé, ce qui est source d'angoisse.

au vécu personnel, familial. Je maintiens ce que j'ai dit en commission : la dignité est inhérente à la condition humaine, et une personne, quel que soit son état physique, voire psychique,

Nos règles particulières font que le scrutin public va permettre de décider massivement de l'adoption ou non de cet amendement. amendement. Il n'est pas exclu que ce vote ne reflète absolument pas la position de cet hémicycle, alors même qu'il est ce matin très fourni. fourni. Je ne sais pas si le groupe qui a demandé un scrutin public entend le maintenir, mais je pense que celui-ci pose un problème. Aussi, je souhaiterais que ce groupe laisse la démocratie se manifester

repose sur la souveraineté populaire, la souveraineté de la Nation, dont nous sommes ici les représentants. C'est le Parlement qui fait la loi et qui décide aujourd'hui de ce qu'il faut faire

qu'il y a quelque chose après la mort, comme ceux qui pensent qu'il n'y a rien ont eu un débat extrêmement noble et respectueux des sentiments religieux et non religieux des uns des autres. Ils ont abordé ces questions en termes de droits.

les expériences qui nous ont été transmises, notamment celle du sénateur Arnaud. En effet, j'ai senti, et je me suis reconnu dans ce qu'il a dit, une longue fréquentation des services de soins palliatifs.

il serait bon que chacun puisse s'exprimer directement par son vote personnel. La liberté de choisir la fin de sa propre vie est un sujet qui touche chacun d'entre nous dans ce qu'il a de plus intime.

L'actualité médiatique vient également nourrir la réflexion et l'émotion collectives par des cas particuliers bouleversants. Il me semble que, à l'instar de nombre de nos voisins européens-

L'allongement de la durée de la vie et le vieillissement de la population rendent chaque jour ce sujet plus prégnant. Je comprends naturellement les réticences des membres du corps médical : mettre fin à une vie heurte profondément le coeur même de leur engagement professionnel et va à l'encontre me semble cependant que les progrès considérables de la médecine, qui se poursuivent et continueront de se poursuivre, nous amènent évidemment à envisager ce débat sous un autre angle. Alors que l'espérance de vie avoisine les 80 ans et que celle des générations qui arrivent aujourd'hui sur cette terre pourrait approcher le siècle, alors que la technologie et le transhumanisme ouvrent des possibilités vertigineuses, je crois qu'il est indispensable d'accepter que toutes et tous ne souhaitent pas poursuivre leur vie dans des conditions de santé ou de forme physique qu'ils jugent insatisfaisantes. Le défi du grand âge, de la maladie et de la détérioration du corps, voire de la conscience, pose cette question avec toujours plus d'acuité.

où la liberté de vote fait qu'ils seront divers. Je trouve très regrettable de ne pas pouvoir voter pour cette loi.

Le scrutin est clos.